La séance est ouverte.

Monsieur le ministre, allons nous laisser le Danemark perdre le Groenland sans rien faire ? Allons nous le laisser seul face aux pressions américaines ? Alors que le roi du Danemark est encore en visite officielle en France, les menaces pesant sur ce vaste territoire autonome sous souveraineté danoise sont plus fortes que jamais end dernier, Donald Trump n’a pas exclu de recourir à la force pour l’annexer ! Certes, le quarante septième président américain nous a habitués à faire des déclarations à l’emporte pièce puis à les oublier, mais il nous a aussi appris que, sous « Trump 2.0 », tout devenait possible ou, à tout le moins, envisageable. La géopolitique est devenue un sous genre de science fiction… Que ferait l’Europe si les États Unis s’emparaient du Groenland ? Rien, évidemment ! Heureusement, ce scénario demeure hautement improbable. En revanche, il est clair que le Groenland est à la croisée des chemins. Dans le monde du dérèglement climatique, le Groenland – un espace grand comme quatre fois la France – devient stratégique, en raison à la fois de sa situation géographique, mais également de ses ressources. Cela n’a pas échappé à la logique de prédation à l’œuvre à la Maison Blanche. Or ce territoire stratégique est un territoire européen ; cela fait deux cents ans qu’il est placé sous souveraineté danoise. C’est aussi un territoire autonome, dont le destin ne dépend que de ses habitants.

Monsieur le ministre, la France compte t elle jouer un rôle actif pour que l’Europe soutienne le Danemark et le Groenland dans cette crise éminemment symptomatique du XXI siècle ? Dans l’affirmative, quelle forme prendrait ce soutien ? La parole

d’un dialogue avec les autorités danoises, de relever leur niveau d’engagement au Groenland. Par ailleurs, contrairement à tout ce que l’on peut lire ou entendre, il n’y a pas d’investissement chinois particulier au Danemark aujourd’hui. Enfin, le Danemark a été exemplaire en annonçant le rehaussement de ses efforts militaires dans la région.

Nos chaînes publiques sont un bien commun, qui contribue au pluralisme et à la diversité culturelle à travers le monde. Mme la ministre affirmait que cette réforme tenait compte des nombreuses consultations des syndicats. Je voudrais bien savoir lesquels ! Ceux qui manifestent depuis 2015 ? Ou ceux qui étaient en grève au cours des deux derniers jours ? Lundi soir, à la Bourse du travail, où ils étaient réunis, leur inquiétude était palpable. Ils craignent d’abord une privatisation à bas bruit, la sous traitance.

les procédures judiciaires concernant des parlementaires, d’anciens présidents, de futures ex candidates, des ministres de l’intérieur ou de la culture… Qui peut leur donner tort ? L’histoire de Canal+ a démontré

un jour près, on aurait pu croire à un poisson d’avril ! Citons quelques extraits des bonnes intentions dont ils se sont fait le serment : il y est question d’une « coopération migratoire confiante, fluide et efficace », de l’« importance de la coopération judiciaire entre les deux pays », de la « confiance dans la clairvoyance du président Tebboune » et d’un appel « à un geste de clémence et d’humanité

Après une série d’incidents diplomatiques et l’humiliation répétée de la France par l’Algérie, comment les Français pourraient ils croire que tout serait réglé, comme par miracle, en un appel téléphonique ?

L’appel qui a eu lieu entre les deux présidents, lundi dernier, a ouvert un espace diplomatique en vue de cette résolution. Cet espace, nous allons nous en saisir,

et indépendants. Monsieur le ministre de l’intérieur, le 4 février dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité, dans un élan transpartisan, la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

je pense bien évidemment au phénomène des mules, qui frappe nos territoires ultramarins, notamment la Guyane, que j’ai l’honneur de représenter dans cet hémicycle. Vous le savez, une grande partie de la cocaïne consommée en France hexagonale et en Europe transite par ces régions. Chaque vol au départ des Antilles ou de la Guyane transporte des mules qui ont ingéré des ovules de cocaïne, au péril de leur vie. Les contrôles renforcés dans les aéroports ont certes permis de ralentir le trafic, mais n’ont pas pu le juguler totalement. De plus, ces contrôles mobilisent quotidiennement les forces de l’ordre, obligées de délaisser d’autres missions, tout aussi essentielles.

nucléaire et de santé doivent délivrer un agrément pour autoriser ces installations, mais la situation est trop grave pour ne pas engager cette démarche au plus vite. Monsieur le ministre, je vous sais préoccupé par ce problème. Je sais que les autorités sont mobilisées et conscientes de l’ampleur du phénomène. Néanmoins, est de constater que plusieurs pays européens se dotent de moyens efficaces pour interpeller les porteurs de boulettes ingérées ou insérées dans leur corps. Alors, pourquoi, malgré la pertinence de cette mesure,

Alors que vous vous apprêtez à signer des décrets engageant notre politique énergétique pour les dix ans à venir, ne pensez vous pas qu’il soit grand temps de tout mettre sur la table, afin de redessiner une réelle stratégie décarbonée et de retrouver l’esprit pionnier d’Edgar Faure ?

Il y a donc, derrière cet enjeu de défossilisation, non pas simplement un enjeu de protection de l’environnement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais un véritable enjeu de souveraineté. En effet, nous ne souhaitons pas

Cette politique, c’est l’ancien monde, celui de l’énergie renouvelable européenne, ce n’est pas du tout le monde de l’énergie décarbonée, dont le nucléaire fait partie. Tout cela coûtera à l’État et aux Français « un pognon de dingue alors que ce budget devrait être employé pour atteindre un seul objectif : l’électrification de nos industries et de nos entreprises. Dès lors, un simple débat ne suffira certainement pas. Il est indispensable de travailler à une véritable loi de programmation sur soixante ans La parole est à M. Bernard Fialaire, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe du RDSE, le plus ancien du Sénat et au nom duquel je m’exprime, a toujours défendu avec ferveur la République, ses valeurs, ses institutions et l’État de droit, fondement de notre démocratie.

produit dans une incandescence médiatique attisée par un vent mauvais, qui souffle de Russie, de Hongrie et même d’une Amérique qui conteste nos valeurs humanistes et progressistes. Héritiers du philosophe Alain, nous défendons le droit et même le devoir de vigilance envers les pouvoirs, tous les pouvoirs, mais notre société a besoin que soient rappelées avec force et conviction les valeurs de notre République. Nous avons besoin de la voix forte et cohérente du Gouvernement, qui incarne aussi ces principes. Nous attendons un discours clair, sans ambiguïté de nos ministres, de tous nos ministres, jusqu’au Premier d’entre eux

Monsieur le ministre, que comptez vous faire pour que l’expression du Gouvernement et le rappel des principes républicains couvrent cette entreprise de dérégulation bien orchestrée, relayée par des médias complices ?

Cette considération circonstancielle de l’autorité judiciaire ne réduit en rien la règle absolue qui s’applique à notre État de droit et à notre démocratie : la séparation des pouvoirs. La justice passe et le Gouvernement ne peut ni commenter ni moins encore contester. Le Parlement seul, s’il le souhaitait, pourrait envisager de modifier la loi qui a conduit à la décision des magistrats. Vous avez cité le philosophe Alain ; je citerai pour ma part Montesquieu : « Les juges de la nation ne sont […] que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres […] qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur. » Au moment où, comme vous l’avez souligné, l’idée même du fonctionnement démocratique fait l’objet de remises en cause à divers degrés dans le monde, nous pensons sage de nous en tenir à ces principes et à leur application.

de remplacement, fragilisées par vos prédécesseurs, ou pour l’école inclusive. Malgré cette volonté affichée, force est de constater que, sur ce dernier point, le compte n’y est pas non plus : les postes d’enseignant demeurent insuffisants pour améliorer significativement le taux d’encadrement, notamment dans le secondaire, ce préalable étant indispensable

à prendre en compte non seulement le taux d’encadrement, qui s’améliorera dans tous les départements, mais aussi le maillage territorial. Je tiens à souligner, madame la sénatrice, qu’il ne peut pas y avoir de fermeture d’école sans l’accord du maire. Si cette règle

j’interrogeais le Gouvernement sur la question douloureuse des expulsions locatives. À l’époque, les mesures de confinement avaient permis le prolongement de la trêve hivernale. L’épidémie de covid 19 étant passée, l’épidémie de misère a repris le dessus : elle continue de toucher de plus en plus de ménages. Pour les ménages plongés dans la précarité, le coût du logement représente jusqu’à 41 % des ressources mensuelles. Le nombre d’impayés de loyers a triplé depuis 2020. En 2024, les expulsions locatives ont augmenté de 87 % par rapport à 2023. est angoissante pour des dizaines de milliers de familles, constituées pour beaucoup de femmes seules avec enfants. Quelque 350 000 personnes sont sans domicile et les centres d’hébergement sont saturés. Notre pays compte pourtant 3 millions de logements vacants, dont 800 000 pourraient être mobilisés immédiatement. 2,7 millions de personnes sont en attente d’un logement, nous savons que nous devrions en construire 200 000 par an. Or les aides publiques à la pierre ont diminué, l’inflation a fait flamber les coûts de la construction et la réduction de loyer de solidarité a asséché les finances des bailleurs publics. publics. Une intervention publique sans précédent s’impose de manière urgente. Quelle politique en faveur du logement pour tous – je dis bien : pour tous – entendez vous mettre en œuvre, madame la ministre ? Comptez vous mettre fin aux expulsions locatives sans relogement, comme l’avait promis en 2017 le Président de la République ?

Nous devons intervenir dès le premier signalement dans le but de réduire le plus possible le recours à la procédure judiciaire d’expulsion. Le budget pour 2025 nous a permis de financer vingt six équipes mobiles dans les territoires les plus en tension. Ces équipes accompagnent les personnes les plus fragiles et éloignées des services sociaux dès la première alerte d’impayés.

la rue en 2023, les niches fiscales relatives au secteur du logement ont coûté près de 11 milliards d’euros aux finances publiques en douze ans. De quoi financer 70 000 logements sociaux ! Madame la ministre, le groupe

ce propos est non pas le mien, mais celui de Florent Menegaux, président du groupe Michelin, devant la commission des affaires économiques du Sénat. Alors que cette entreprise emploie 132 000 personnes en Auvergne, en France et dans le monde entier,

je sais aussi que le budget des transports vient de subir une coupe claire de plusieurs millions d’euros. Les 4 millions d’habitants des onze départements du Massif central sont isolés. Sur une carte de France isochrone, Clermont Ferrand, seule métropole française non desservie par le TGV, est relégué au même rang que la Côte d’Azur, à trois heures

Face à ce constat désastreux en matière de mobilité, les gueux des volcans d’Auvergne attendent une forte volonté politique de désenclavement et d’aménagement du territoire. Monsieur le ministre, comment comptez vous faire fonctionner normalement la ligne Paris Clermont

Pour y remédier, l’État a engagé des moyens importants : plus de 365 millions d’euros ont été investis dans les nouvelles rames et près de 900 millions d’euros dans la régénération et la modernisation du réseau. Monsieur le sénateur,

C’est pourquoi – cela ne vous aura pas échappé, monsieur le sénateur, car vous l’avez rappelé – j’ai fait de ce dossier l’une de mes priorités. J’ai eu l’occasion de vous rencontrer deux fois sur ce sujet dans le cadre d’un groupe de travail transpartisan

j’emprunterai évidemment cette ligne ! – afin d’y tenir un comité de suivi des dessertes ferroviaires et d’évoquer à l’intention des différentes parties prenantes, notamment des usagers, des propositions et des mesures concrètes de court, de moyen et de long terme. Surtout, monsieur le sénateur Boyer, j’espère vous redonner enfin l’envie de prendre le train ! La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Il s’agit d’une véritable ingérence dans la vie des entreprises françaises. Elle relève de la croisade mondiale que les États Unis entendent mener contre l’égalité entre les femmes et les hommes, l’inclusion des travailleurs handicapés et la lutte contre les discriminations

Quelle initiative comptez vous prendre pour que l’Union européenne porte la parole de la France et défende des valeurs qui sont aussi les siennes ? Pour conclure par un sujet dans le sujet, comment le Gouvernement entend il protéger les salariés français des entreprises américaines

Rossignol, nous avons en effet pris connaissance de plusieurs courriers transmis par l’administration américaine – je dis bien l’administration américaine dans son ensemble – l’ambassade à un certain nombre d’entreprises françaises, leur enjoignant de « mettre fin à la discrimination illégale » et de « rétablir les opportunités […] basées sur le mérite ». que ces courriers ne reflètent que les valeurs du gouvernement américain. Ce ne sont pas les nôtres ! Cette pratique n’est pas acceptable. Je regrette profondément ces lettres. Elles ne sont à la hauteur ni de l’amitié séculaire entre nos deux pays et nos deux peuples ni du partenariat qui nous lie.

Le Président de la République a pris l’initiative, avec le Premier ministre et le Gouvernement, de réunir les filières concernées à l’Élysée jeudi prochain. Nous dialoguerons avec nos entreprises afin de leur apporter le secours que vous proposez Le temps me manque pour développer tous ces sujets, mais soyez certaine que le Gouvernement sera à leurs côtés dans ce qui est malheureusement une bataille, que j’espère provisoire. Ainsi, nous serons solidaires, unis et efficaces pour défendre ces valeurs. La

en réaction, a lancé une enquête antidumping sur les importations de brandy et de cognac venant d’Europe, qui a conduit à soumettre ces produits à des droits de douane de 35 %. Nous venons d’apprendre que l’application définitive de droits de douane supplémentaires est reportée au 5 juillet

En choisissant la voie réglementaire, le Gouvernement ne fait qu’appliquer l’article L. 141 1 du code de l’énergie. Ce qui est juridiquement irréprochable l’est moins philosophiquement : ce décret n’est pas anodin. En l’occurrence, le décret fixant la troisième PPE, qui doit couvrir la période 2025 2035, est stratégique pour atteindre la neutralité carbone, mais il va au delà. De notre planification énergétique dépend la France de demain. Ce document doit refléter une vision et une ambition nationales que nous avons jusqu’ici peiné à avoir. Toutes majorités confondues, nous n’avons agi que par lois successives, sans vue d’ensemble. Des choix purement politiciens ont été faits, de Fessenheim et du projet Astrid. Nous nous sommes perdus dans des querelles stériles pour ou contre le nucléaire et les énergies renouvelables (EnR). La stratégie énergétique dont nous avons besoin est indissociable de notre volonté de réindustrialiser et de réarmer. C’est l’œuf et la poule : sans énergie, pas d’industrie ni de réarmement, et inversement., de notre vision énergétique dépendent la souveraineté, la puissance et la prospérité de demain. De tels choix engagent toute la Nation. Monsieur le ministre, pourquoi vous passez vous de l’expertise du Sénat ?

Cette suppression sera sans doute confirmée en séance publique la semaine prochaine. Je rappelle que ces restrictions ont pour origine une directive européenne de 2008 prise sur le fondement d’une alerte de l’Organisation mondiale de la santé, laquelle évaluait alors à 47 000 le nombre de décès

des critères inadaptés ou encore l’absence d’offre de mobilités substitutives et d’accompagnement de l’État. Ce texte avait été précédé d’un rapport de l’Assemblée nationale et a été suivi d’une mission créée par Élisabeth Borne, alors Première ministre. Les conclusions et recommandations de ces deux rapports sont proches et font état d’une mise en œuvre défaillante, qui exclut des cœurs de ville les populations les plus fragiles, ce qui pose des problèmes d’équité et donc d’acceptabilité. Dans ce contexte,

D’une conférence nationale sur l’eau, version « Michel Barnier », à des conférences régionales, version « François Bayrou », quelle est la méthode de travail ? Quel rôle le Comité national de l’eau jouera t il ? Qu’en sera t il des comités de bassin ?

Tout cela est bien faible au regard des besoins ! Deux ans après les annonces du plan Eau, moins de 5 % des aires de captage sont protégées. Personne n’est dupe : nous reportons toujours à demain le traitement des urgences du moment. Madame la ministre, la politique de l’eau reste t elle une priorité de votre ministère ?

remercie de votre question et de votre engagement sur le sujet de l’eau. Je pense en particulier à votre rapport d’information publié en 2023, qui a beaucoup enrichi nos réflexions. Nous fêtons aujourd’hui, quasiment jour pour jour, les deux ans du plan Eau, qui avait été lancé le 30 mars 2023 par le Président de la République et par mon prédécesseur Christophe Béchu.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la situation dans les Balkans. Dire qu’elle est préoccupante serait un doux euphémisme… La Bosnie Herzégovine fait face aux velléités de sécession de Milorad Dodik à la tête de la Republika Srpska. La Serbie connaît d’importantes manifestations et une crise politique qui perdure. Le Kosovo est toujours sous tension ethnique. La Macédoine du Nord, elle, est confrontée à la colère de sa jeunesse. Telle est la triste situation des Balkans occidentaux aujourd’hui, monsieur le ministre – vous ne la connaissez que trop bien. Alors que la guerre russo ukrainienne persiste, les pays balkaniques traversent une grave crise dont personne ne semble pouvoir pronostiquer l’issue.

ci, par son instabilité politique, devient une proie facile pour des ingérences anti européennes. La France et l’Union européenne y ont des attaches fortes et anciennes, un rôle diplomatique à jouer et des intérêts à défendre.

jour pour jour la guerre faisait rage dans cette région, au cœur de l’Europe. Vous l’avez dit, en Serbie, les autorités font face à une contestation populaire sans équivalent dans l’histoire récente.

à la suite du verdict prononcé à son encontre, le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, multiplie les initiatives et les mesures sécessionnistes, que nous avons toutes fortement dénoncées. Nous avons donné notre accord pour un renforcement de l’opération Eufor Althea, mission sous commandement français – c’est le général Cottereau qui la commande. Une force de réserve intermédiaire sera prête à intervenir en cas de dégradation de la situation sécuritaire. Elle a été déployée le 16 mars dernier, 400 personnels supplémentaires Le ministre délégué Benjamin Haddad se rendra demain à Sarajevo afin de poursuivre les échanges avec les autorités centrales et de rencontrer les représentants des partis d’opposition de Republika Srpska.

le 16 mai prochain se tiendra à Tirana, en Albanie, le sommet de la Communauté politique européenne. Ce sera l’occasion pour le Président de la République d’échanger avec l’ensemble des chefs d’État et de gouvernement des pays concernés. Pour conclure, madame

: il s’agit à la fois de permettre à chaque jeune de bâtir sa voie de réussite et de nous doter des compétences dont notre pays aura besoin demain. Vous l’avez rappelé, depuis 2018, cette compétence est partagée entre l’État et les régions, l’État étant chargé de l’éducation et de l’orientation et les régions de l’information sur les métiers. Dans le même temps, de nombreux dispositifs ont été mis en place pour permettre aux élèves d’élargir leurs horizons et de faire des choix éclairés. Je pense notamment à la découverte des métiers dès le collège, au stage de seconde, au développement de dispositifs tels que les cordées de la réussite, ou encore à la création d’un bureau des entreprises

débouche souvent sur du décrochage. Et l’on ne saurait ignorer que le monde économique a besoin de compétences, pour ce qui est notamment des métiers d’avenir. J’ai naturellement poursuivi les concertations qui avaient été engagées notamment par ma prédécesseure et par le ministre Portier. De nombreuses contributions ont été présentées, par les organisations patronales, par les régions, par les collectivités en général. La synthèse est en cours et je suis évidemment à l’écoute,

Imaginez un pays où le parti arrivé en tête lors de deux élections nationales successives se voit privé du pouvoir par les vaincus du suffrage universel. Quatre millions d’euros ! Imaginez un pays où la première chaîne de télévision, critique du pouvoir, est fermée d’office.

Cette décision ne vise pas seulement une femme politique : elle frappe la figure majeure de l’opposition, celle qui a rassemblé des millions de Français et qui incarne la principale alternative à votre gouvernement. Rendez l’argent ! Il ne s’agit de rien d’autre que d’une tentative inacceptable d’écarter une adversaire politique par des moyens qui n’ont plus rien à voir cela le droit ! Nous sommes, au Sénat, les garants des droits et des libertés. Mes chers collègues, qu’importe nos différences – et elles sont nombreuses –, vous le savez tous : le droit d’interjeter appel est un droit fondamental, indissociable de la présomption d’innocence. Ce que nous vivons aujourd’hui en France, c’est l’application des méthodes d’un régime autoritaire : une justice instrumentalisée qui frappe l’opposition au moment même où cette dernière menace le pouvoir. Vous condamnez les pires dictatures, mais un pays où le droit au recours est bafoué n’est plus un État de droit. Quand un dirigeant autoritaire condamne un opposant, vous dénoncez l’autoritarisme. Et quand cela se produit en France, il n’y aurait là qu’une simple affaire judiciaire ? Qui peut croire que cette décision n’est pas un coup porté à la liberté du peuple français de choisir ses représentants ? Ne nous y trompons pas : si aujourd’hui vous souhaitez affaiblir Marine Le Pen,… Elle s’affaiblit toute seule ! … demain d’autres figures de l’opposition subiront le même sort. Ce précédent ouvre la voie à un régime où le pouvoir en place choisit ses adversaires et dicte les termes du débat démocratique. Monsieur le Premier ministre, comment garantiriez vous l’indépendance des magistrats quand plus d’un tiers d’entre eux font allégeance au Syndicat de la magistrature, celui là même qui a appelé en juin dernier à se mobiliser contre l’accession au pouvoir de ce qu’ils appellent l’« extrême droite

veut dire que la séparation des pouvoirs doit être respectée. Vous ne pouvez pas prétendre que la justice serait instrumentalisée ou aux mains du Gouvernement, pas plus que vous ne pouvez contester une décision de justice. La seule initiative que le Parlement est susceptible de prendre, c’est de faire évoluer la loi en vertu de laquelle cette décision de justice a été rendue. Mais, pour avoir été parlementaire à l’époque

! Je me tiens donc rigoureusement à la position qui est et restera celle du Gouvernement : nous ne commentons ni ne contestons aucune décision de justice

Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle figurera dans l’analyse politique du scrutin concerné. J’informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anticriminalité organisée,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

Madame la présidente, madame la présidente de la commission économiques, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, qu’il vous appartient d’examiner aujourd’hui, rejoint une priorité du Gouvernement : lutter contre la fraude partout où elle se trouve et faire payer à chacun ce qu’il doit à notre société. Cette proposition de loi est le fruit du travail de mon prédécesseur, Thomas Cazenave. Qu’il me soit donc permis, avant toute

mais également lorsqu’elle a trait aux aides publiques, car elle porte préjudice à nos concitoyens, à nos finances publiques, à la confiance que les citoyens portent à l’État et,, au contrat républicain qui nous lie tous. Nous sommes déterminés à renforcer les moyens juridiques permettant de traquer et de punir tous types de fraudes. Ce que nous avons accompli en matière de lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière, nous devons le réaliser aussi en ce qui concerne la fraude aux aides publiques.

Nous allons poursuivre ces avancées dès cette année en maintenant les ressources allouées à la lutte contre la fraude fiscale et en renforçant les moyens budgétaires attribués à Tracfin. Nous nous attaquons également, avec Catherine Vautrin, Astrid Panosyan Bouvet et Yannick Neuder, à la fraude sociale et à la fraude médicale. La solidarité à la source déployée le mois dernier, qui permet désormais le préremplissage des déclarations mensuelles de ressources pour les allocataires du revenu de solidarité active améliorera la fiabilité des calculs, contribuera à réduire les fraudes et facilitera la vie des honnêtes gens. Il me semble que c’est une bonne solution pour avancer. Nous poursuivrons également le déploiement de 1 000 agents supplémentaires chargés de la lutte contre la fraude sociale jusqu’en 2027 au sein des caisses du régime général et nous investirons 1 milliard d’euros d’ici à 2027 pour moderniser les systèmes d’information, qui sont des éléments désormais indispensables à la détection et à la punition de la fraude. la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, nous avions prévu de renforcer l’échange des données entre l’assurance maladie et les complémentaires santé, tout en poursuivant la sécurisation de la carte Vitale.

loin. Ces chiffres, mesdames, messieurs les sénateurs, ne sont pas que des statistiques abstraites ou désincarnées. Je l’affirme clairement : le drame de la fraude, c’est aussi qu’elle finance l’industrie du crime organisé. J’ai eu l’occasion récemment de remercier nos douaniers pour leur engagement inébranlable et leur bilan exceptionnel, notamment en matière de lutte contre le narcotrafic. En 2024, nous avons saisi 111 tonnes de stupéfiants sur le territoire national pour une valeur de 1,2 milliard également démantelé quatre vingt douze réseaux criminels. Au delà de la saisie des biens et de la drogue, c’est bien au portefeuille que nous devons frapper les criminels afin de les asphyxier financièrement. Ce constat fonde l’action des services de Bercy contre le blanchiment et la fraude financière. Il justifie aujourd’hui la nécessité de lutter contre la fraude aux aides publiques qui profitent à ces réseaux.

Les fraudes liées au certificat d’économies d’énergie (C2E) ou encore celles qui sont liées à MaPrimeRénov’ ont causé des préjudices de plusieurs centaines de millions d’euros en 2023. Une partie de ces fonds a été retrouvée transférée à l’étranger grâce aux détections de Tracfin. Si nous n’agissons pas, ces pratiques frauduleuses sont vouées à se développer, à aggraver encore davantage le déficit de nos finances publiques et à altérer la confiance de nos concitoyens à l’égard de l’État. Il est donc aujourd’hui impératif d’agir avec force, détermination et efficacité. C’est pourquoi la discussion qui s’ouvre aujourd’hui sur cette proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques est absolument déterminante pour garantir la capacité de l’État à protéger les citoyens, à mener les politiques publiques efficaces et à préserver ses finances.

Vous avez notamment véritablement permis d’accentuer le mécanisme général de lutte contre la fraude à la source, qui permet de suspendre ou de rejeter une aide publique dès lors qu’il existe des indices sérieux de fraude.

Le texte vise également à améliorer la coordination entre les administrations publiques pour renforcer leurs prérogatives, en particulier dans les cas de suspicion de fraude à une aide publique.

J’en profite pour saluer le travail important de la mission interministérielle de coordination antifraude (Micaf), qui est un rouage essentiel de cette coordination entre les administrations. En ce qui concerne les En ce qui concerne les prérogatives des administrations, vous avez également voulu renforcer les conditions du contrôle et la sanction. Vous avez ainsi accru les pouvoirs de sanction de la DGCCRF et les pouvoirs de contrôle des inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Plusieurs mesures ont été prises pour accroître les contrôles, protéger les bénéficiaires, obliger à la transparence concernant les prestations des sous traitants ou renforcer l’interdiction du démarchage abusif. À cet

À cet égard, le délai de conservation des photos et des vidéos dans le cadre du contrôle par horodatage et géolocalisation en matière de C2E est désormais fixé à six ans, contre cinq ans initialement. Je conclurai, mesdames, messieurs les sénateurs, en vous disant qu’il est logique que ceux qui financent le crime organisé soient criminalisés. Jusqu’à maintenant, voler son voisin en bande organisée était un acte criminel,

Il faut que nous fassions preuve de cohérence dans les sanctions que nous appliquons à ceux qui fraudent, qu’ils fraudent ou qu’ils volent leurs voisins, ou qu’ils fraudent ou qu’ils volent l’État. Ainsi, ce texte, vous le voyez, s’inscrit dans notre ambition de lutter contre toutes les fraudes de doter l’administration de tous les moyens juridiques nécessaires, dans le plein respect de notre État de droit, pour combattre efficacement ceux qui volent l’État et les Français.

la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à lutter contre la fraude aux aides publiques, principalement dans les domaines de la rénovation et de l’efficacité énergétiques. En effet, ces secteurs sont particulièrement sujets aux montages frauduleux : en 2023, la rénovation énergétique est le deuxième secteur le plus pourvoyeur de signalements sur SignalConso, la plateforme de réclamation de la DGCCRF. Je me réjouis que ce texte ait reçu un accueil particulièrement favorable au sein de la commission des affaires économiques. Je remercie notre présidente, Dominique Estrosi Sassone, de m’avoir confié cette mission, qui me tient à cœur. Vous connaissez ici mon engagement acharné en faveur de la simplification des normes, au sein notamment de la délégation sénatoriale aux entreprises. Je remercie également le rapporteur pour avis, Antoine Lefèvre, du travail qu’il a accompli sur les articles délégués au fond à la commission des finances. Je pense que nous avons cherché, lui comme moi, à améliorer le texte, en vue de renforcer l’efficacité du dispositif de lutte antifraude et la protection du consommateur. Le texte de la commission a selon moi trois objectifs proposer des choses simples, éviter la surréglementation et permettre à nos administrations d’effectuer un saut qualitatif dans la lutte contre la fraude. fraude. Aujourd’hui, nos administrations sont dimensionnées pour arrêter le fraudeur qui conduit à 140 kilomètres à l’heure sur l’autoroute, mais pas celui qui roule à 200 kilomètres à l’heure et fait des blessés Pour mieux armer toutes les administrations face aux fraudeurs, l’article 1 de la proposition de loi introduit un pouvoir de suspension pendant trois mois de l’instruction d’une aide publique en cas de suspicion de fraude, sur le modèle de ce qui est déjà applicable en matière sociale. Ce pouvoir de suspension sécurisera leurs décisions face aux recours contentieux. Notre commission l’a conforté en permettant que cette suspension soit renouvelée une fois, afin de donner un temps suffisant aux agents pour infirmer ou confirmer la fraude. Je dirai ensuite un mot du démarchage téléphonique. Les députés ont en effet introduit, au sein du présent texte, l’article 1 de la proposition de loi de notre collègue Pierre Jean Verzelen pour un démarchage téléphonique consenti et une adoptée à l’unanimité par le Sénat le 14 novembre dernier. C’est la preuve qu’il existe une volonté politique partagée de tous bords d’avancer rapidement dans la lutte contre ce phénomène qui exaspère les Français. S’il convient de saisir l’occasion de cette proposition de loi sur laquelle est engagée la procédure accélérée, nous soulignerons jusqu’au bout l’origine sénatoriale de ce dispositif. C’est pourquoi j’émettrai un avis favorable sur les amendements de notre collègue Pierre Jean Verzelen, qui visent à reprendre sa proposition de loi, au delà de son seul article 1. Il a tenu aussi à introduire certains dispositifs consensuels adoptés par les députés : je salue son esprit de responsabilité et de dialogue. En revanche, alors que nous avons adopté à l’unanimité sa proposition de loi le 14 novembre dernier, je constate que nombre d’entre nous souhaitent revenir sur ce consensus en introduisant des exceptions. Je le regrette, car chaque exception ouvre la voie à d’autres et fragilise le texte dans son ensemble, les contrôles comme la compréhension du dispositif par les consommateurs. En outre, je souligne que nous n’empêcherons pas les entreprises de faire leur travail en appelant leurs clients : le texte vise bien à prévoir une « exception client » qu’il n’est pas question de remettre en cause. Gardons en tête l’objectif, qui est de donner du répit aux consommateurs face à des appels intempestifs, qui nous exaspèrent tous ! Outre le démarchage téléphonique, cette proposition de loi vise à interdire la prospection commerciale par voie électronique dans les secteurs de la rénovation énergétique et de l’adaptation des logements. Cela concerne les messages personnels de prospection par SMS, e mails ou encore par messages sur les réseaux sociaux. Je précise, car c’est important, qu’il ne s’agit en aucun cas d’interdire la publicité ou la communication des entreprises sur les réseaux sociaux, qui resteront possibles. Seuls sont visés les messages personnels. Nous souhaitons simplement limiter l’effet de report du démarchage téléphonique abusif vers le démarchage électronique. Dans le secteur de la rénovation énergétique, où le démarchage téléphonique est interdit depuis 2020, les entreprises malhonnêtes se rabattent sur les messages électroniques, dont nous sommes de plus en plus inondés. J’insiste donc sur l’intérêt de préserver cette mesure. Pour protéger le consommateur face aux comportements frauduleux d’entreprises, l’article 3 renforce l’information du consommateur concernant la sous traitance et la détention de labels conditionnant l’accès à des aides publiques, comme le label Reconnu garant de l’environnement (RGE), qui est indispensable pour bénéficier de MaPrimeRénov’. de l’importance des montants financiers en jeu pour les ménages, il est crucial qu’ils aient bien en tête ce que la sous traitance peut impliquer en termes d’éligibilité aux aides publiques. La commission a donc renforcé le dispositif, en tenant compte des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique de 2023. Elle a étendu les cas dans lesquels la DGCCRF peut suspendre le label RGE ou l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’ et a introduit un délai de carence durant lequel l’entreprise frauduleuse ne peut pas recandidater à un label. De manière plus générale, la commission a renforcé les pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, ainsi que les suites à donner à ses enquêtes. Parce que le travail en silo est l’ennemi de la lutte contre la fraude, la commission a accru les échanges d’informations entre la DGCCRF, l’Ademe, l’Anah et les organismes de qualification des entreprises réalisant les travaux ou les organismes de certification des diagnostiqueurs. Dans d’autres domaines, nous avons également renforcé les échanges d’informations entre la DGCCRF et le ministère de la justice, par exemple. la commission a adopté un amendement visant à renforcer encore davantage les contrôles et les sanctions en matière de certificats d’économies d’énergie.

Quant aux sanctions, vingt sont publiées chaque année au ; elles ont conduit à des annulations, pour 20 millions d’euros, et à des amendes, pour 9 millions d’euros. On mesure tout le chemin qu’il reste à parcourir pour passer du contrôle à la sanction ! En outre, à l’article 5, la commission a sécurisé le dispositif de contrôles visuels à distance (CVAD) des C2E. Enfin, la commission a introduit un article 6 visant à faciliter l’échange d’informations entre la Commission de régulation de l’énergie et la DGGCCRF, à la demande de ces organismes. Elle a également ajouté un article 8 tendant à faciliter le contrôle à distance des fraudes aux compteurs communicants par Enedis et GRDF, cette disposition convenant à ces acteurs, ainsi qu’à la CRE et au médiateur national de l’énergie Je vous proposerai, quant à moi, trois amendements. L’un d’eux vise à élargir l’accès à l’Observatoire DPE Audits. Les deux autres sont purement rédactionnels. Nous aurons l’occasion d’en débattre. sont, mes chers collègues, les apports de la commission des affaires économiques à cette proposition de loi contre les fraudes aux aides publiques, que je vous invite à adopter largement. Très bien

Dans un contexte de hausse de la fraude, en particulier aux aides à la rénovation énergétique, il était nécessaire d’agir. Le texte que nous examinons aujourd’hui constitue l’aboutissement de travaux menés par notre collègue député Thomas Cazenave lorsqu’il était ministre des comptes publics. Je suis bien conscient que ce texte ne constitue pas le Grand Soir de la lutte contre la fraude aux aides publiques. Ah ! Cependant, il contient plusieurs mesures intéressantes à cet égard, qui permettront – je l’espère – de faciliter le travail des services enquêteurs et d’enrayer les comportements frauduleux. Les articles délégués au fond à la commission des finances sont les articles 2 à 2 , 3 C, 3 et 3 . Je présenterai par conséquent la position de la commission sur ces mesures. D’abord, plusieurs dispositions assez consensuelles visent à faciliter l’échange d’informations entre acteurs de la lutte contre la fraude. Il en va ainsi de l’article 2, qui prévoit notamment une clause générale permettant à l’ensemble des administrations d’échanger librement des informations en cas de suspicion de fraude, et plus spécifiquement aux agents préfectoraux de recevoir des informations des organismes de protection sociale. De même, l’article 2 vise à faciliter l’accès des agents de l’Agence de services et de paiement (ASP) au fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba). Les articles 2 et 2 visent, enfin, à renforcer les moyens d’enquête de Tracfin et de l’inspection générale des finances, grâce à l’extension de leur droit de communication. Je suis favorable à l’adoption de ces articles, qui ont connu, pour certains, des améliorations légistiques et de fond lors de l’examen du texte en commission. J’en viens maintenant aux articles 3 et 3 , qui prévoient des mesures d’encadrement de la sous traitance sur le marché des travaux de rénovation. Ces articles ont suscité beaucoup de débats lors de leur examen par la commission des finances. L’article 3 limite à deux rangs le nombre de sous traitants pour la réalisation de travaux ouvrant droit à certaines aides à la rénovation énergétique telles que MaPrimeRénov’. L’article 3 , vise, quant à lui, à étendre cette limitation aux travaux ouvrant droit à MaPrimeAdapt’. La commission s’est montrée favorable à cette mesure, qui apporte une réponse aux risques de fraudes qu’implique la sous traitance en cascade. L’article 3 prévoit également une obligation pour l’entreprise qui facture des travaux de rénovation énergétique de disposer du label Reconnu garant de l’environnement pour qu’un projet soit éligible aux aides publiques. Je précise que cette qualification, qui permet de garantir la qualité et la durabilité des travaux de rénovation, n’est aujourd’hui obligatoire que pour les entreprises qui réalisent effectivement ces travaux. Il faut bien le reconnaître, cette disposition concerne davantage la structuration du marché de la rénovation énergétique que la lutte contre la fraude. Toutefois, la commission des finances s’est positionnée en faveur de cette mesure. L’obligation de qualification RGE pour l’entreprise donneuse d’ordre présente en effet un certain intérêt puisqu’elle permet de limiter l’émergence sur le marché de la rénovation énergétique de sociétés opportunistes, qui sous traitent des marchés à des entreprises RGE tout en ne disposant elles mêmes d’aucune qualification. J’avais toutefois alerté la commission des finances sur les risques qu’impliquerait l’introduction immédiate de cette disposition dans notre droit. Je souhaite réitérer cette mise en garde devant notre assemblée. Une adoption précipitée de cette disposition aurait un effet néfaste sur l’offre de travaux de rénovation puisqu’elle conduirait à exclure du marché un certain nombre d’acteurs dont le modèle ne permet pas de disposer du label RGE. Je pense, notamment, aux grandes enseignes de bricolage. Il ressort de mes auditions qu’elles ne présentent pas de risque particulier de fraude. Or elles proposent des parcours de travaux dont la qualité semble reconnue par les consommateurs. Il ne me semble pas opportun d’utiliser le prétexte de la lutte contre la fraude pour évincer ces acteurs du marché alors que, dans le même temps, les pouvoirs publics encouragent une politique ambitieuse d’incitation de nos concitoyens à rénover leurs logements. Dans un esprit de compromis, la commission des finances a donc proposé de décaler la date d’entrée en vigueur de cette disposition au 1 janvier 2027 afin de laisser au Gouvernement le temps de définir des critères de qualification pour ces entreprises par voie réglementaire. Sans anticiper les débats que nous aurons tout à l’heure dans l’hémicycle, je relève que le Gouvernement propose de repousser l’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions des articles 3 et 3 au 1 janvier 2028. Madame la ministre, comme je viens de le démontrer, je partage votre préoccupation sur l’importance de ne pas précipiter l’application de ces mesures afin d’éviter de déstabiliser le marché de la rénovation.

En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement, je demande, au nom de la commission des affaires économiques, que l’examen de l’article 3 et des amendements portant articles additionnels après l’article 3 soit réservé après l’examen de l’article 3,

Madame la ministre, il faut écouter le Sénat et les parlementaires. Il est nécessaire de changer de logiciel : arrêtons d’ouvrir les robinets et de contrôler après.

d’effacer l’amende fiscale du groupe Vivendi de 320 millions d’euros, malgré des erreurs délibérées dans les comptes, envoie un message délétère et renforce l’impunité des délinquants en col blanc.

climatique ne pourront pas être atteints. Lundi dernier encore, la ministre de la transition écologique annonçait pourtant vouloir conjuguer écologie et amélioration du quotidien des Français, en prônant une écologie « populaire Elle a insisté sur la nécessité de renforcer notre souveraineté, de soutenir l’industrie française et de rendre la transition énergétique accessible à tous. Nous partageons cet alors, comment justifier la baisse des crédits octroyés à la rénovation énergétique ? Comment expliquer que, dans le même temps, le budget de MaPrimeRénov’ soit amputé de 500 millions d’euros ? Si nous voulons réellement aider les ménages à rénover leurs logements, réduire notre dépendance énergétique et soutenir le secteur de la construction locale, alors il faut des moyens concrets, et pas seulement des déclarations Je le rappelle, le secteur du bâtiment représente environ 45 % de la consommation d’énergie et près de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Plus de 5 millions de logements sont encore considérés comme des passoires thermiques. Pourquoi Parce que nous devons correctement hiérarchiser les problèmes. La transition écologique est prioritaire et la lutte légitime et nécessaire contre la fraude ne doit pas devenir un paravent.

C’est inconstitutionnel, et vous le savez. D’autre part, si l’on veut lutter contre la fraude sociale, il faut encourager la déclaration plutôt que le travail clandestin. Ainsi, sur les 1,6 milliard d’euros de fraudes

les obligations des plateformes numériques de déclarer et de prélever les cotisations des microentrepreneurs. Bref, il faut un texte solide sur ce sujet et ne pas fragiliser par des cavaliers législatifs la faible ambition de cette proposition de loi de lutter contre la fraude aux aides énergétiques. Le deuxième débat concerne le niveau de sous traitance autorisé. Il faut raccourcir les circuits et mieux contrôler les responsabilités. Oui, autoriser deux rangs de sous traitance est progrès passer à trois serait un recul. Enfin, le dernier débat porte sur l’évaluation de l’efficience des travaux, et donc des aides. Pour nous, c’est simple : celui qui facture doit être celui qui fait le devis. Si n’importe quelle entreprise commerciale – on a parlé de magasins physiques, mais

contre les fraudes aux aides publiques, adoptée à l’Assemblée nationale en janvier dernier. En introduction, je souhaite mettre l’accent sur un phénomène qui se développe, à savoir le recours aux propositions de loi alors que les textes émanent visiblement de l’exécutif. Rappelons que le premier signataire de ce texte est Thomas

à la protection du consommateur et à la lutte contre la fraude aux aides publiques : c’est un impératif pour renforcer le consentement à l’impôt de nos concitoyens. Dans le temps qui m’est imparti, j’aborderai certaines dispositions parmi les plus notables de cette proposition les articles examinés au fond par la commission des affaires économiques. J’évoquerai aussi quelques uns des amendements de notre groupe. Je laisserai ma collègue Isabelle Briquet aborder les articles examinés pour avis par la commission des finances. Ce texte permet ainsi de suspendre temporairement l’octroi ou le versement d’une aide publique en cas d’indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré. de rejeter expressément l’octroi ou le versement d’une aide lorsque la fraude est avérée. Je salue l’apport des députés socialistes sur ces points, qui ont sécurisé le dispositif juridique en précisant que les indices doivent être « sérieux », notion déjà consacrée par la jurisprudence.

à l’augmentation du taux de pénalité appliqué à la somme à rembourser lorsque le bénéficiaire de l’aide l’a obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes. Des dispositions de cette proposition de loi visent à lutter contre la fraude aux la fraude aux travaux de rénovation énergétique et d’adaptation à la perte d’autonomie avec des dispositions interdisant le démarchage, des obligations d’information relatives à la sous traitance et à la détention du label RGE. Je défendrai des amendements tendant à interdire le démarchage à domicile dans le domaine de la rénovation énergétique, énergétique, afin de mieux protéger les consommateurs concernés, souvent âgés. Le renforcement de la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie est un axe fort de cette proposition de loi. Le texte sécurise l’action du Pôle national des certificats d’économies d’énergie lors de ses contrôles, facilite la détection de fraudes lors de l’instruction des demandes de C2E et renforce la sanction que le Pôle peut prononcer. Nous sommes favorables au renforcement du partage d’informations entre la DGCCRF et la Commission de régulation de l’énergie afin de mieux lutter contre la recrudescence de la fraude fiscale dans le secteur de l’énergie. De même, nous approuvons les mesures qui renforcent les échanges de données entre la DGCCRF, l’Ademe, l’Anah, les organismes de qualification et le ministère de la justice. de conforter les missions de la DGCCRF, mais il faut renforcer ses moyens humains, en particulier pour lutter contre la fraude à MaPrimeRénov’ : tel est l’objet d’un de nos amendements. J’approuve également le renforcement de la constatation des fraudes commises sur les compteurs communicants, renforcement très attendu par Enedis, GRDF, la CRE et le médiateur national de l’énergie. Nous proposerons un amendement visant à renforcer juridiquement le dispositif.

madame la ministre, mes chers collègues, les sénateurs du Rassemblement national accueillent avec bienveillance cette proposition de loi qui permet de mieux s’équiper pour mener la chasse aux fraudeurs. La fraude est un véritable fléau et constitue une trahison du contrat social. Compte tenu de la situation économique du pays provoquée par huit années de macronisme, la lutte contre les fraudes aux aides publiques et contre toutes sortes de fraudes doit devenir une priorité nationale pour redresser les finances publiques : c’est un enjeu de justice. Si nous voulons réellement faire des économies et renforcer la confiance des Français dans les politiques publiques, il est impératif de tendre vers la tolérance zéro face aux fraudeurs. Chaque euro fraudé est en effet un euro volé aux honnêtes Français. Permettez moi de rappeler quelques chiffres de la Cour des comptes, qui illustrent l’ampleur du problème : la fraude aux aides publiques, c’est environ 1,5 milliard d’euros par an ; la fraude sociale, près de 15 milliards d’euros ; la fraude fiscale, entre 30 milliards et L’Insee, pour sa part, estime que la fraude à la TVA représente un manque à gagner pour l’État de plus de 20 milliards d’euros. Ces chiffres sont alarmants au vu de notre situation budgétaire. Ces milliards d’euros pourraient profiter aux honnêtes Français, mais, une fois de plus, ce sont les citoyens respectueux des règles qui sont pénalisés ou qui subissent des restrictions injustes. Il est donc impératif de démanteler les réseaux de la fraude organisée qui détournent les aides publiques destinées aux entreprises françaises. Ces réseaux mafieux fragilisent les dispositifs mis à disposition des entrepreneurs. Afin de lutter efficacement contre ces pratiques, il est nécessaire de durcir les dispositifs en vigueur. Cela passe d’abord par un renforcement des contrôles, grâce à des moyens humains et technologiques adaptés, puis par une simplification des procédures pour détecter plus rapidement les anomalies et diminuer les zones d’ombre favorables aux fraudeurs, enfin par des sanctions dissuasives et adaptées à la gravité des infractions. Seule la création d’un ministère consacré à la lutte contre toutes les formes de fraudes pourra nous permettre de mener la chasse aux fraudeurs de manière efficace, comme le préconisait Marine Le Pen dans son programme présidentiel. Une structure ministérielle dédiée, avec un parquet unique qui centralise les plaintes de fraudes, serait en mesure de coordonner les efforts entre les différentes administrations, de centraliser les données et de garantir une traque efficace des fraudeurs. Mes chers collègues, cette proposition de loi marque un premier pas important dans la lutte contre la fraude, la fraude pénalisant toujours les bons élèves. En s’attaquant aux abus qui coûtent chaque année des milliards d’euros à l’État, le texte traduit la volonté politique de protéger les ressources publiques et de rétablir la justice sociale. Notre groupe soutient cette initiative, convaincu qu’elle répond aux attentes des citoyens. Cependant, pour qu’elle porte ses fruits,

La proposition de loi doit être le point de départ d’une stratégie ambitieuse et cohérente visant à restaurer la confiance dans nos institutions et non un simple coup de com’ destiné à donner l’impression que l’on apporte des solutions au problème majeur que constitue la fraude.

en quittant le ministère des comptes publics, en septembre dernier, Thomas Cazenave a emporté dans ses cartons ses projets pour lutter contre la fraude. Redevenu parlementaire, trois semaines plus tard, il déposait sur le bureau de l’Assemblée nationale sa proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques. Après son examen par les députés au mois de janvier, le texte nous est présenté aujourd’hui. Cette proposition de loi est utile et nécessaire.

Chaque euro d’aide publique indûment versé est un euro qui manquera à nos écoles, à notre armée, à nos hôpitaux, à notre police, à notre justice – dont on parle tant –, à nos caisses de retraite… Je m’arrête là Comme élus, et dans nos permanences, nous avons les uns et les autres constaté les attentes grandissantes en matière de travaux de rénovation et d’isolation thermique. Qui n’a pas été sollicité pour un dossier MaPrimeRénov’ qui prenait trop de temps

Les fraudeurs font peser sur les professionnels une suspicion généralisée. Cette proposition de loi vise à permettre aux artisans honnêtes, qui sont l’immense majorité, de s’appuyer sur ces dispositifs publics pour travailler et développer Ce texte va également permettre à nos administrations, notamment Tracfin, de mieux détecter les fraudes grâce à un partage d’informations renforcé. Les moyens d’action de la DGCCRF et de l’inspection générale des finances seront renforcés. Il leur sera désormais permis d’accéder à des documents jusqu’ici couverts par le secret professionnel. Si la proposition de loi est adoptée, le versement des aides publiques pourra être temporairement suspendu J’en viens à un point qui a déjà été abordé et qui me tient à cœur : le démarchage téléphonique. Si cela ne vous ennuie pas, mes chers collègues, je résumerai ce qui s’est passé ces derniers mois.

Le texte Cazenave est débattu en commission à l’Assemblée nationale au mois de janvier et la députée Delphine Batho propose un amendement visant

efficacité et à bon escient. Lorsqu’il y a fraude, le contrat est incontestablement remis en cause. C’est alors la crédibilité de l’action publique qui est en jeu.

la possibilité de suspendre temporairement le versement d’une aide publique en cas de suspicion sérieuse de fraude. En second lieu, il renforce la coopération entre les services de l’État et facilite le partage d’informations entre les administrations afin de mieux détecter

sujet crucial pour notre pacte social et nos finances publiques. En mai 2023, le ministre chargé des comptes publics a lancé un plan de lutte contre les fraudes sociales, fiscales et douanières,

100 équivalents temps plein seront redéployés pour le contrôle douanier du e commerce. Enfin, plus de 1 milliard d’euros seront alloués à la modernisation des outils numériques de détection.

Le travail doit être néanmoins poursuivi et amplifié. Le contrôle de certaines aides publiques pourrait en effet être amélioré, notamment celui des certificats d’économies d’énergie. Dans un

Enfin, nous proposons de rappeler l’obligation pour les employeurs et les organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, de dresser la liste des parties autorisées à échanger librement les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions et de prévoir un système d’information partagé et dématérialisé. Mes chers collègues, mieux lutter contre la fraude aux aides publiques, c’est préserver la confiance de nos concitoyens dans l’action publique. En effet, les aides publiques sont un pilier de notre pacte social. Elles permettent d’accompagner des initiatives économiques, de soutenir les plus vulnérables et d’encourager la transition écologique.

ma grand mère, sage paysanne bretonne,

pour les organisations criminelles qui détournent les aides publiques en réalisant des montages de sociétés, ces dispositifs constituent une véritable manne financière.

s’engagent pourtant dans une démarche vertueuse, mais coûteuse, de rénovation qui subissent les conséquences les plus lourdes de ces pratiques frauduleuses. Ces fraudes sont enfin insupportables dans le contexte de raréfaction des ressources publiques. Alors que chaque euro d’argent public doit compter, chaque comportement frauduleux est une injure lancée à l’ensemble des acteurs, publics ou privés, qui rationalisent au mieux leurs budgets, leurs subventions, qui vont chercher coûte que coûte l’efficience, malgré le contexte économique très difficile. Il est donc grand temps de mieux contrôler l’utilisation de l’argent du contribuable et de protéger davantage le consommateur. Il est grand temps de rénover nos dispositifs antifraudes afin que le panel des aides à la rénovation ressemble un peu moins au Far West.

d’activité. Sans compter les millions d’euros qui nous échappent… Cette fraude silencieuse et insidieuse, qui infiltre nos dispositifs comme un poison lent, poursuit son œuvre à l’ombre des radars. présente proposition de loi constitue une avancée, mais elle demeure insuffisante face à l’ampleur du problème. Nous ne pouvons plus nous contenter de pansements pour stopper l’hémorragie financière causée par une fraude systémique et organisée. Nous avons industrialisé la dépense ; il est vital d’industrialiser le contrôle, en le dotant d’une colonne vertébrale robuste et agile. En premier lieu, avant de multiplier les dispositifs d’aides et autres chèques, encore faudrait il s’assurer que les conditions de contrôle et d’évaluation soient réunies et opérationnelles.

En second lieu, nous devons œuvrer à briser les silos administratifs qui entravent l’efficacité de notre action. La création en 2020 de la mission interministérielle de coordination antifraude a été un premier pas,

et non des pincettes. Enfin, la transparence doit être au cœur de notre démarche. Les citoyens doivent retrouver la confiance. S’ils acceptent l’effort fiscal, ils doivent être assurés que celui ci ne sert à nourrir ni les parasites ni les fantômes administratifs. égard, la création d’un fichier national des fraudeurs contribuerait à atteindre cet objectif. Mes chers collègues, agissons avec courage, volonté politique et détermination pour plus de justice sociale, en envoyant d’urgence un signal fort à ceux qui fraudent, mais aussi à ceux qui paient : les contribuables, les collectivités, les entreprises

la proposition de loi déposée par l’ancien ministre chargé des comptes publics Thomas Cazenave s’attaque à un sujet important : la fraude aux aides publiques. Celle ci se manifeste sous différentes formes falsification de pièces justificatives, présentation de fausses informations, surfacturation de travaux ou prestations fictives, recours abusif à la sous traitance, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique. Le secteur de la rénovation énergétique est particulièrement touché. Les dispositifs comme MaPrimeRénov’ ou les certificats d’économies d’énergie sont devenus des cibles privilégiées pour les fraudeurs. En 2023, la fraude aux C2E a représenté un manque à gagner de 480 millions d’euros pour l’État, tandis que les mouvements suspects liés à MaPrimeRénov’ s’élevaient à 400 millions d’euros.

Je m’attarderai à présent sur l’article 3, réécrit en commission par le rapporteur, qui affaiblit le dispositif voté par l’Assemblée nationale concernant la sous traitance dans le secteur de la rénovation énergétique. En l’état, cet article garantit l’effectivité du dispositif encadrant la sous traitance en cascade pour bénéficier de MaPrimeRénov’ et de l’éco PTZ. Il reporte également à 2027 l’obligation pour l’entreprise facturant les travaux de disposer du label Reconnu garant de l’environnement. tel report ne me semble pas opportun. Cet article passe en revanche sous silence le problème majeur des fraudes aux C2E. Celles sont souvent le fait d’entreprises commerciales opportunistes, qui utilisent des montages opaques de sous traitance pour capter les aides publiques sans garantir la qualité des travaux. Il ne s’agit pas ici de remettre en cause l’activité des enseignes de bricolage, mais il est légitime de s’assurer que les aides bénéficient en priorité aux entreprises qualifiées et compétentes et non à des structures commerciales, dont l’unique objectif est de capter les aides publiques. Lorsqu’il s’agit de fonds publics, nous devons être intransigeants : seuls les professionnels certifiés doivent pouvoir bénéficier des aides. Par ailleurs, si la lutte contre la fraude sociale et la fraude aux aides publiques est nécessaire, je déplore que la fraude fiscale soit trop souvent laissée dans l’ombre. Le manque à gagner lié à la fraude fiscale oscille pourtant entre 80 milliards et 100 milliards d’euros par an.

L’asymétrie entre le traitement politique de la fraude sociale et celui de la fraude fiscale est difficilement justifiable sur le plan moral et économique. Il est légitime de sanctionner les abus liés aux aides publiques, mais cette rigueur doit s’appliquer également aux fraudes massives dans le domaine fiscal.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, si la rénovation énergétique est un levier essentiel pour améliorer la performance de nos logements et atteindre nos objectifs climatiques, elle ne doit certainement pas devenir une opportunité pour les fraudeurs. C’est tout l’enjeu de cette proposition de loi, qui tend à renforcer les contrôles et les sanctions pour garantir que les fonds publics bénéficient bien à ceux qui en ont réellement besoin. Chaque année, les fraudes aux aides à la rénovation coûtent des centaines de millions d’euros à l’État. Ce détournement d’argent public mine la confiance des Français, pénalise les citoyens honnêtes et prive les ménages les plus modestes d’un soutien financier indispensable. Ce texte, très attendu par les professionnels du secteur, est d’autant plus nécessaire que la fraude prend plusieurs formes : entreprises malveillantes facturant des travaux inutiles, bâclés ou inexistants, sociétés frauduleuses montant des dossiers au nom de particuliers à leur insu,

des anomalies ont été relevées dans 51 % des entreprises contrôlées. Ce phénomène, dont l’ampleur exacte reste difficile à mesurer, doit être combattu avec des outils à la hauteur des enjeux. Madame la ministre, nous rencontrons fréquemment sur le terrain des entrepreneurs, des artisans et des maîtres d’œuvre

– c’est indispensable –, afin de laisser aux administrations le temps nécessaire de mener des enquêtes approfondies et de garantir que les fonds publics ne soient pas détournés. Garantir la limitation de la sous traitance en cascade à deux rangs

tel encadrement garantirait la qualité des travaux, limiterait les fraudes et assurerait que les aides publiques profitent réellement aux ménages et aux professionnels qualifiés. Nous reviendrons sur ce sujet Si cette proposition de loi vise à répondre à un grand nombre de problématiques, il est également essentiel de s’attaquer à un autre frein majeur : la complexité administrative des aides à la rénovation énergétique. Critères d’éligibilité flous, dossiers rejetés à cause d’erreurs mineures, délais de versement trop longs

manifestement, ce texte ne sera pas le grand soir de la lutte contre la fraude, mais il va dans le bon sens. Dans le même esprit, on ne voit pas bien pourquoi l’on y a fait figurer une réforme des règles du démarchage commercial, mais, là aussi, cette nouvelle réglementation va globalement dans le bon sens.

Chaque année, des milliards d’euros d’aides publiques sont mobilisés pour soutenir notre économie, accompagner nos entreprises, protéger les plus fragiles et préparer l’avenir. Ce sont nos impôts, notre argent, notre confiance collective qui sont investis dans ces dispositifs. Malheureusement, une part de ces aides est détournée par des fraudeurs organisés. À n’en pas douter, certaines de ces fraudes pourraient, demain, être prévenues par une plus grande célérité de l’administration dans sa réaction lorsqu’elle suspecte une fraude. Actuellement, les administrations disposent de moyens limités pour agir face à des soupçons de fraude lors de l’instruction d’une demande d’aide publique. Grâce aux dispositions de l’article 1, les agents habilités pourront suspendre, pour une durée initiale de trois mois, l’octroi ou le versement d’une aide publique quand ils sont en présence d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquements délibérés. Cette suspension, renouvelable une fois, leur offrira le temps nécessaire pour mener des investigations approfondies, tout en préservant les droits des demandeurs de bonne foi. En revanche,

de son pouvoir de suspension, le cas échéant comme moyen de procéder, en fin d’exercice surtout, à des réductions budgétaires. On l’a vu par le passé ! Les ministres devront donc, au moyen de circulaires, préciser et harmoniser les critères de suspension, mais aussi rappeler que les décisions de suspension, outre qu’elles devront toujours être suffisamment motivées, pourront dans tous les cas faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.

Verzelen pour cette initiative, qui induit un changement fondamental et attendu dans la réglementation du démarchage téléphonique. Le système, en vigueur depuis 2016, de la liste d’opposition dite Bloctel va disparaître au profit d’un régime généralisé de consentement préalable du consommateur à recevoir régime bien plus protecteur de sa vie privée et de son bien être. Ce nouveau cadre légal, couplé à la possibilité d’infliger des sanctions sévères, doit nous inciter à produire un texte équilibré, c’est à dire à la fois protecteur des intérêts des consommateurs et attentif au maintien et au développement d’une prospection commerciale respectueuse des lois et des bonnes pratiques. Il ne faut en aucun cas pénaliser des secteurs économiques entiers du fait de quelques acteurs délinquants ; la tranquillité de nos concitoyens, mais aussi la préservation des entreprises et des emplois concernés doivent être notre boussole.

à limiter les effets pervers que pourrait avoir un allongement de la durée de suspension des aides publiques, en conditionnant la prolongation de ce délai à la réalisation d’investigations dans le délai initial de trois mois.

il faut avoir à l’esprit que les investigations sont menées au bénéfice du pétitionnaire. Cela signifie que, si au terme du délai,

vise à faire en sorte que les demandes d’octroi d’une aide publique ayant fait l’objet d’une mesure de suspension et pour lesquelles la suspicion de fraude a été levée puissent être examinées prioritairement. Quel est l’avis de la commission

quelle que soit leur origine, même frauduleuse, pouvaient entrer dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel. Ainsi, les dettes tenant à un versement indu de RSA pourraient être examinées dans le cadre d’une procédure de surendettement, donc effacées. À l’inverse, les sommes indûment versées par les organismes de protection sociale en sont toujours exclues, et ce au détriment d’une certaine logique. La précision ainsi opérée par le Conseil d’État crée une insécurité pour les départements, qui pourraient se voir refuser le recouvrement des créances de RSA frauduleuses du fait de leur possible effacement à l’occasion d’une procédure de surendettement. Bien que cette possibilité d’effacement de dette ne soit pas systématique, les magistrats devant juger de la bonne foi du requérant, il apparaît inéquitable que les dettes de RSA exigibles du fait ne puissent pas bénéficier du même régime de protection que les prestations versées par les organismes de protection sociale à l’égard des procédures de surendettement des particuliers.

Ce n’est pas un simple détail technique ; c’est une exigence de notre État de droit. La Cour de cassation elle même, dans un arrêt du 22 septembre 2021, rappelle que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée aux buts poursuivis. Autrement dit, s’il peut y avoir atteinte à la vie privée, cette atteinte doit rester encadrée, justifiée et surtout contrôlée. Seul le juge est à même d’exercer ce contrôle. Lui seul peut en effet apprécier si l’information sollicitée est véritablement indispensable ou si d’autres voies moins intrusives auraient pu être explorées.

selon lequel les garanties démocratiques constitueraient des obstacles et la justice serait un frein à l’action publique. Nous ne pouvons l’accepter. Notre position est simple : oui, les échanges d’informations entre administrations doivent être facilités lorsque cela est nécessaire à la conduite de l’action publique, mais, non, cette efficacité ne saurait se faire au prix de nos principes fondamentaux. Garantir le contrôle du juge, ce n’est pas entraver les enquêtes, c’est les légitimer, c’est prévenir les abus, c’est préserver la confiance des citoyens en nos institutions. La parole est à M. Gérard Lahellec,

Le fichier relatif aux données de réservation des passagers aériens, dit PNR, est autorisé par la loi à titre expérimental et a été mis en œuvre à l’issue d’un travail approfondi de la Cnil. Il est accessible aux agents des ministères de l’intérieur, de la défense et des transports, ainsi qu’à ceux des douanes pour les besoins liés à la prévention de certaines infractions qui concernent les actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Cette création à titre expérimental, protégée par de nombreux garde fous, se comprend au vu de la sensibilité des informations qui y sont contenues. La liberté d’aller et de venir doit être protégée. Par conséquent, il ne me semble pas possible d’adopter cet amendement. Il conviendrait, pour opérer une modification aussi ample que celle proposée, de consulter la Cnil en amont. Il serait en outre nécessaire, ce que cet amendement n’a pas pour objet de prévoir, de modifier les dispositions du code de la sécurité intérieure afin d’éviter de créer une incompatibilité entre les différents codes. je ne nie pas que la fraude sociale pourrait diminuer largement grâce à un accès au PNR. En effet, cet accès faciliterait la détection de faux résidents français. J’invite donc le Gouvernement à avancer sur le sujet. Pour toutes ces raisons,

dans la mesure où les données API PNR sont collectées par les compagnies aériennes pour des finalités précises – prévention et constatation des actes de terrorisme ; prévention et constatation des infractions pour lesquelles un mandat d’arrêt pour atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État est exigé –, qui ne comprennent pas la lutte contre la fraude sociale.

de cet amendement part d’une exigence simple, mais fondamentale, celle de la clarté républicaine. Cette proposition de loi consacrée à la lutte contre la fraude est particulièrement nécessaire, elle ne saurait servir de prétexte à des insinuations plutôt dangereuses. L’alinéa 15 que nous proposons de supprimer établit un lien à peine voilé entre immigration et fraude. Ce lien est fallacieux et – disons le clairement – choquant. est fallacieux, parce qu’aucune donnée sérieuse ne permet d’étayer une quelconque corrélation structurelle entre l’origine des personnes et leur propension à frauder. La fraude est un acte, pas une identité. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur lui même a reconnu le caractère problématique de cette rédaction et a proposé une réécriture de l’alinéa, qui n’a pas été retenue. Nous le regrettons, mais il n’est peut être pas trop tard pour corriger le tir

d’ajout – je dirai même de dérive. Surtout, cette disposition constitue une atteinte à la protection des données personnelles des usagers. Habiliter les agents des services préfectoraux à accéder à des données sociales, y compris sensibles, quelquefois sur la base de simples soupçons

L’adoption des amendements identiques n 20, 70 et 113 viendrait faire échec à la mise en œuvre de la réciproque de ce que dispose actuellement l’article L. le deuxième alinéa dudit article établit que les agents des services préfectoraux habilités peuvent transmettre les renseignements utiles à la lutte contre la fraude sociale aux organismes de protection sociale, l’inverse n’est pas prévu aujourd’hui. Étant favorable

la construction européenne. Cependant, de nombreuses évolutions ont été mises en œuvre pour lutter contre la fraude sociale transfrontalière. Depuis le mois de juin 2023, le système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (Eessi) fonctionne et permet un échange sécurisé d’informations dans un cadre conforme à la réglementation. Il relie 3 400 organismes des 32 pays participants : les 27 États membres de l’Union européenne, auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse et le Royaume Uni. Par conséquent, cet amendement est satisfait par l’existence de ce type d’échanges.

de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale toute information utile pour contrôler l’ouverture des droits et le montant des prestations, recouvrer des créances ou vérifier les conditions de délivrance de documents d’entrée et de séjour sur le territoire national. Par conséquent, ils participent

fond, la discussion que nous aurons à l’article 8.

à la rénovation énergétique ou dans des carrousels de TVA. Néanmoins, le dispositif proposé me paraît peu opérant. Il revient à introduire des soupçons à l’égard d’entrepreneurs sur le fondement de signaux faibles, dont aucun ne révèle en lui même une pratique illégale.

HCFiPS que vous avez cité, le code de la sécurité sociale autorise déjà, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, les agents chargés du contrôle à mener leur investigation au profit de plusieurs organismes. Par exemple, si les contrôleurs de la caisse des allocations familiales constatent l’absence d’un allocataire sur le pour l’ensemble des risques. Comme l’indique le rapport, le problème est donc moins législatif que relatif au manque de publicité de ce dispositif, qui n’est pas toujours identifié par les caisses. J’invite donc le Gouvernement à appuyer la démarche interne nécessaire pour faire connaître le droit existant au sein de la direction de la sécurité sociale.

impôts. La transmission des documents par voie postale et sous format papier n’est plus adaptée aux modalités de communication actuelles. C’est pourquoi cet amendement vise à imposer que les réponses au droit de communication bancaire prennent désormais la forme de flux dématérialisés.

Les agents de la DGFiP et les services douaniers chargés de la lutte contre les fraudes doivent pouvoir disposer d’informations facilement exploitables dans le cadre de leurs contrôles. La dématérialisation des informations transmises me semble d’autant plus importante

pour obtenir ces informations, ce qui engendre des délais importants et mobilise inutilement des ressources administratives. Nous proposons donc de moderniser l’accès à ces données en supprimant cette contrainte procédurale. Quel est l’avis de la commission des finances ?

Comme pour l’Agence de services et de paiement, cet amendement vise simplement à automatiser et à rendre plus fluide un échange d’informations qui existe déjà. En outre, sa rédaction dispose que les informations transmises doivent être nécessaires aux missions d’enquête et de contrôle. Cela permet d’assurer la proportionnalité du dispositif. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

notamment en cas de non respect par les professionnels des injonctions de mise en conformité, lorsque ceux ci manquent à leurs obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Beaucoup des fraudes que nous observons sont fortement entremêlées avec des réseaux de criminalité organisée, y compris le narcotrafic.

des finances, concerne le droit de communication des membres de l’inspection générale des finances, laquelle exerce une double compétence : le contrôle des organismes publics et parapublics, ainsi qu’un rôle de conseil auprès du Gouvernement.

de faux documents pour obtenir indûment des fonds publics. L’administration pourrait ainsi refuser une nouvelle déclaration pendant quatre ans en cas de fraude avérée et pendant cinq ans si les sommes indûment perçues ne sont pas remboursées. Ce levier est essentiel pour protéger les fonds publics destinés

révélant des indices sérieux de fraude ou d’opposition à un contrôle. Une suspension pour une durée maximale de quatre mois limiterait le versement de fonds publics à ces structures, en attente de la décision définitive de l’État. Elle inciterait également les organismes à coopérer pleinement

les fraudes aux aides publiques, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique. Toutefois, encore faut il que les moyens suivent. Il nous semble ainsi nécessaire de vérifier, pour les renforcer le cas échéant, que les moyens humains de la

contrôles en matière de formation professionnelle en clarifiant les règles de communication des informations et en solidifiant le système d’échange dématérialisé entre les acteurs concernés. Actuellement, l’absence de coordination entre les services de l’État, les financeurs et les certificateurs limite la détection rapide des fraudes, qui sont pourtant en forte augmentation. En permettant un partage horizontal des alertes et une meilleure programmation des contrôles, nous renforcerions la lutte contre les fraudes

sur la qualité de la formation professionnelle a mis en évidence, en octobre 2023, un développement important de la fraude aux différents dispositifs d’aide à la formation professionnelle. Nous avons tous en tête les nombreux cas de fraude au compte personnel de formation. Dans ce contexte, il me semble

contrôle du décret d’application de la loi par la Cnil. Par ailleurs, la question de l’efficacité d’une telle mesure se pose. Les organisations criminelles utilisant de fausses adresses pourraient évoluer simplement en utilisant des adresses existantes tenues par des hommes de paille. Enfin, l’incidence des développements informatiques nécessaires pour donner cet accès dans de bonnes conditions n’a pas été évaluée.

d’abord, l’amendement du rapporteur affaiblit les avancées votées à l’Assemblée nationale. Il revient sur l’interdiction faite aux entreprises non qualifiées RGE de sous traiter des travaux, en renvoyant à un décret d’application et en repoussant l’entrée en vigueur de la

En outre, l’article 3 reste silencieux sur les certificats d’économies d’énergie, pourtant eux aussi largement concernés par des pratiques frauduleuses. Il est urgent de fermer la porte aux sociétés opportunistes, souvent créées à la seule fin de capter des aides publiques au moyen de démarchages agressifs et de fausses promesses. L’enjeu est non pas de pointer tel ou tel acteur du marché, mais bien de faire preuve de clarté sur le type de sociétés qui posent problème : des structures commerciales sans qualification qui n’ont accès à ces aides que grâce à la possibilité de sous traiter à des artisans RGE. Tant que cette faille subsistera, la fraude

Nous pensions qu’il était nécessaire de créer un dispositif de qualité pour les entreprises qui réalisent la facturation auprès des particuliers. D’où ce délai. Toutefois, je vous annonce d’ores et déjà que

Ce sujet a déjà été largement débattu en commission et, sur le fond des dispositions, je souscris à la réécriture de l’article que propose le Gouvernement. L’extension du champ d’application de l’article à l’ensemble des travaux de rénovation énergétique aidés me semble bienvenue. Il s’agit d’éviter de créer des distorsions entre les différents types de travaux selon les aides auxquelles ils ouvrent droit. L’assouplissement à trois rangs du nombre de sous traitants pour les travaux qui concernent plusieurs logements au sein d’un même bâtiment me semble également pertinent. La limitation à deux rangs de sous traitants est en effet trop restrictive dans certains cas de figure. Toutefois, comme je le disais tout à l’heure, la date d’entrée en vigueur au 1 janvier 2028 proposée par le Gouvernement n’est pas assez ambitieuse. Je vous rejoins, madame la ministre, pour considérer qu’une entrée en vigueur immédiate aurait un impact négatif sur l’offre de travaux de rénovation à court terme. Elle pourrait déstabiliser certaines entreprises dont le modèle d’affaires repose sur le recours à plusieurs sous traitants et qui, dans la grande majorité des cas, n’adoptent pas de comportements frauduleux. Sur cette partie de l’article, une date d’entrée en vigueur au 1 janvier 2026 semble néanmoins suffisante pour laisser le temps à la filière de se réorganiser. C’est ce que je propose au travers de mon sous amendement. Concernant la disposition relative à l’obligation de labellisation des entreprises réalisant la facturation des travaux aidés, je préconise d’en rester à la position d’équilibre adoptée par la commission des finances : la date d’entrée en vigueur du 1 janvier 2027 laissait au Gouvernement le temps de définir des critères de qualification. À l’inverse, je Gouvernement le temps de définir des critères de qualification. À l’inverse, je suis défavorable aux initiatives de certains collègues visant à fixer l’entrée en vigueur de l’obligation de labellisation pour les entreprises qui réalisent de la facturation au 1 janvier 2026. La création de critères de qualification nécessitera un certain temps.

pour les entreprises qui ne peuvent disposer d’un tel label actuellement. Nous avons beaucoup parlé des entreprises de bricolage, mais nous aurions pu évoquer les entreprises générales de construction à rayonnement local, qui ne sont pas qualifiées RGE et qui sous traitent les lots de travaux aidés. Il s’agit de s’assurer que ces acteurs puissent continuer à exercer sur le marché de la rénovation énergétique, tout en respectant un certain niveau de qualification. Il ne me semble pas opportun d’utiliser cette proposition de loi pour les évincer purement et simplement du marché. Au risque de me répéter, j’estime que le Gouvernement doit disposer de suffisamment de temps pour consulter les acteurs concernés et définir des critères de qualification sur mesure. Une mise en œuvre précipitée de ce dispositif aurait un effet néfaste sur l’offre de travaux de rénovation à court terme. Une entrée en vigueur au 1 janvier prochain serait prématurée. Cette échéance ne permettrait pas d’élaborer ces textes d’application dans de bonnes conditions.

les trois rangs de sous traitance sont rapidement atteints. Paradoxalement, mes chers collègues, l’adoption de vos sous amendements pourrait même,, encourager la concentration du marché, en favorisant les gros opérateurs intégrés et polyvalents, au détriment des TPE PME et des artisans. Je demande donc le retrait de ces sous amendements, qui sont contraires à la position de la commission

est ainsi rédigé. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie ce jour, sont consultables sur le site du Sénat. En l’absence d’observations, je les considère comme adoptées.